l'ANCOLS, qui est la structure contrôlant les HLM, s'est d'une certaine façon autosaisie pour modifier les règles

présenter l'amendement n° II-211 rectifié. Le présent amendement vise à adapter le dispositif voté par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition du Gouvernement, consistant à créer une mesure d'incitation fiscale pour les travaux de rénovation de logements situés dans nos coeurs de ville. Nos centres-villes anciens comprennent en effet de nombreux immeubles qui ont été ou sont encore affectés à des activités tertiaires, comme des bureaux, des locaux d'associations ou d'administrations, et dont l'état ne permet plus aujourd'hui, ou dans de très mauvaises conditions, d'y exercer ces activités. La transformation de ces bâtiments en logements doit contribuer à la revitalisation de nos centres-villes. Elle ne pourra être effective qu'à la condition de bénéficier de la réduction d'impôt mise en place par le Gouvernement. La parole est à Mme Valérie Létard,

excellente loi votée très majoritairement non seulement par l'Assemblée nationale, mais aussi par le Sénat de la République par 213 voix contre 123 si mes souvenirs sont exacts, le Gouvernement a fait

des opérations de revitalisation des territoires. Ces ORT doivent permettre de « booster » la rénovation, non seulement dans les 222 villes du programme « Action coeur de ville », mais aussi dans l'ensemble de ces villes

être transformés en logements, ce qui contribuerait de manière très forte à la redynamisation de ces territoires. Tel est l'objectif de cet amendement, qui va tout à fait dans le sens des dispositions votées par le Parlement.

prévoit un mécanisme anti-inflationniste, qui empêche le coût du dispositif de croître d'une année sur l'autre- il ne peut évoluer, le cas échéant, qu'à la baisse -, l'enjeu

quand vous faites une revue du zonage, vous avez toujours des perdants et toujours cette même contrainte. Aujourd'hui, j'émettrai un avis défavorable sur ces amendements pour la raison suivante : nous nous sommes engagés à lancer une expérimentation dans la région Bretagne.

Le Gouvernement propose d'instaurer une aide fiscale pour inciter les particuliers à acquérir et à rénover des logements en vue de les louer. L'objectif est d'intervenir sur la dégradation du parc privé des centres-villes. Les travaux devront représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. L'acquéreur doit s'engager à louer le logement ainsi rénové pour une durée comprise entre six et douze ans. Il est proposé d'appliquer cette mesure dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, la liste de ces communes étant fixée par arrêté, et dans les communes s'inscrivant dans un projet global de territoire ayant signé une convention dans le cadre des opérations droit à une réduction d'impôt, calculée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que le dispositif Pinel d'aide à l'investissement locatif. Le champ de la mesure nous paraît trop restrictif. Celle-ci risque de ne pas s'appliquer aux communes rurales, qui ont pourtant besoin de dispositifs incitatifs pour redonner de l'attractivité à leur centre. Elles se retrouvent souvent privées de tout soutien public car elles ne sont couvertes

pour présenter l'amendement n° II-211 rectifié. Le présent amendement vise à adapter le dispositif voté par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition du Gouvernement, consistant à créer une mesure d'incitation fiscale pour les travaux de rénovation de logements situés dans nos coeurs de ville. Si l'on peut se féliciter de la mise en place d'un tel dispositif pour réhabiliter l'habitat ancien, la limitation du prix de revient à 300 000 euros pour le calcul de la réduction d'impôt mésestime le coût important des travaux à entreprendre pour réhabiliter l'habitat ancien dans les centres-villes. Cet habitat est souvent très dégradé- les chantiers coûtent extrêmement cher -, inadapté aux attentes actuelles de nos concitoyens et non respectueux des normes environnementales.

400 000 euros, dans des zones où,, le marché du logement n'est pas particulièrement tendu ! La somme commence à être relativement importante.

Ce nouveau dispositif permettra à un investisseur prêt à s'engager sur douze ans de location de bénéficier, pendant toute cette durée, d'une réduction d'impôt de 21 % du programme, plafonnée à 300 000 euros, dont 2 % l'an pendant les neuf premières années, la réduction d'impôt maximale annuelle pouvant ainsi atteindre 6 000 euros. Cette réduction d'impôt viendra, selon la règle commune, s'ajouter aux autres réductions d'impôt dont l'investisseur pourrait bénéficier- pour emploi à domicile ou au titre d'autres réductions récurrentes pour des opérations réalisées dans le passé -dans le calcul du plafond des réductions d'impôt de 10 000 euros.

monsieur le président. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à supprimer le dispositif introduit par la loi de finances pour 2018, sur l'initiative de la commission des finances, qui limite le montant des frais et commissions directes et indirectes ouvrant droit à la réduction d'impôt Pinel. Nous ne sommes pas favorables à cette suppression.

Au-delà des apparences, le budget de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », ou AGTE, reconduit les moyens de cette mission sur la trajectoire qui était la sienne l'an dernier et qui, en réalité, est la sienne depuis bien des années. Vous ne vous étonnerez donc pas que je sois amené à reconduire mes observations en en accentuant encore un peu la tonalité critique, non par plaisir de critiquer, mais parce que nous sentons bien que nous tutoyons de plus en plus une certaine ligne jaune, couleur décidément à la mode. Sur les crédits de la mission consacrés au financement de la vie politique, le programme 232, l'enveloppe destinée aux partis politiques restera stabilisée en 2019. Il est cependant à noter qu'une somme de l'ordre de 2 millions d'euros ne sera pas dépensée, qui correspond à la pénalité pour défaut de parité. Je recommande au Gouvernement de consacrer cette somme à la politique en faveur des femmes. Je dirai un mot sur la Commission nationale des comptes de campagne. Ses attributions et ses moyens ont été augmentés. Elle peut recourir à des experts pour apprécier les conditions dans lesquelles sont facturées des prestations de service aux candidats. Cet apport est utile si nous ne voulons pas que le contrôle des comptes par cette instance paraisse trop léger et laisse place finalement à des phases judiciaires plus systématiques encore qu'aujourd'hui. Venons-en maintenant à nos territoires. Une fois encore, le réseau préfectoral devra rendre des emplois, comme il l'a fait dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'État, ou RéATE, mais cette fois en dehors de tout cadrage de ces économies d'effectifs, sinon celui qui est inscrit dans la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Mission non prioritaire, mission seconde sinon secondaire, année après année, le réseau d'administration générale de l'État se dévitalise aux dépens des territoires ruraux. Le nombre des sous-préfectures réduites à l'état de simple apparence ne cesse de s'accroître. De 58 en 2017, le nombre de sous-préfectures disposant de moins de 10 emplois passe à 76 en 2018. Cet étiolement, qui touche particulièrement le monde rural, conduit à s'interroger sur les évolutions qu'il pourrait préfigurer. Quels sont vos projets, monsieur le ministre, pour la représentation de l'État au niveau des arrondissements ? Il est vrai que, désormais, les sous-préfectures n'offrent plus d'accès de proximité aux Français depuis la fermeture des guichets du réseau préfectoral. C'était la composante majeure du plan Préfectures nouvelle génération que de s'appuyer sur la numérisation d'un certain nombre de procédures pour supprimer 1 300 emplois et en redéployer 2 700 vers les missions retenues comme prioritaires lutte contre la fraude aux titres sécurisés, contrôle de légalité, ingénierie territoriale et animation des politiques publiques gouvernementales. Cette dématérialisation des procédures s'est traduite par une formidable restriction de l'accès aux services offerts, mais aussi par des difficultés très sérieuses pour obtenir la délivrance de certains titres. Il y a, vous le savez, un problème majeur avec les cartes grises, qui handicape lourdement nos concitoyens. Je relève au passage que la plupart des cartes grises sont aujourd'hui délivrées en dehors de l'intervention de vos services, parfois pour un surcoût illégitime sur lequel il conviendrait d'être particulièrement vigilant. Je rappelle d'ailleurs que le Défenseur des droits recommande d'offrir une solution de remplacement aux demandes dématérialisées pour les nombreux Français qui n'ont tout simplement pas accès à ce moyen. Emplois supprimés, donc, mais, pour ce qui est des emplois redéployés, il faudra patienter. S'agissant de l'animation des politiques publiques et de l'ingénierie territoriale, c'est à une crise que nous avons affaire. Le Gouvernement réfléchit à une réorganisation de l'État territorial : quels éléments pouvez-vous nous livrer sur la prise en compte des difficultés rencontrées par la coordination des services de l'État par les préfets et du nécessaire renforcement de la valeur ajoutée par ces services pour nos territoires ? Envisagez-vous, monsieur le ministre, de créer une administration territoriale de l'État spécifique, comme vous y a engagé le rapport CAP 2022 ? Quelles améliorations de positionnement et de missions entendez-vous apporter à la déconcentration administrative ? J'aurais souhaité finir sur une note plus positive en relevant l'effort réalisé en 2018 pour mettre à niveau certaines capacités d'accueil des étrangers en France. Il n'était que temps. Cependant, il reste encore à faire. Monsieur le ministre, nous vous demandons de veiller à ce que les dépenses de contentieux soient enfin maîtrisées, tant pour celles qui résultent des responsabilités de l'État que pour celles qui résultent du fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant, qui, au vu de certaines conditions d'accomplissement de la mission verbalisatrice, nous paraît comporter quelques risques de dérapage. Moyennant ces observations, mes chers collègues, la commission des finances vous propose d'adopter les crédits de la mission «

programme qui rassemble, à l'exception du programme 333, cette année encore- ce sera modifié l'année prochaine -, les moyens des préfectures, sous-préfectures et représentations de l'État dans les collectivités d'outre-mer, des moyens de nouveau de nouveau en baisse, comme on le sait. Ainsi le schéma d'emploi pour 2019 prévoit-il la suppression de 200 équivalents temps plein, Pour l'administration territoriale, les années et les réformes « ambitieuses » se suivent, accompagnées du même refrain : faire plus et répondre à l'attente de proximité des citoyens usagers avec des moyens en personnels de plus en plus réduits, par la magie de la numérisation, de la mutualisation et de l'externalisation des tâches. À se demander si la meilleure administration n'est pas celle qui se passe de fonctionnaires et d'agents publics Le plan Préfectures nouvelle génération, ou PPNG, était censé permettre de moderniser la délivrance des titres, tout en supprimant 1 300 emplois.

Pendant plusieurs mois, les démarches des usagers ont été fortement perturbées en raison de dysfonctionnements techniques des systèmes informatiques dédiés à ces titres. À ces dysfonctionnements techniques sont venus s'ajouter les effets d'un manque de clairvoyance quant à la réception par les usagers des procédures de dématérialisation des démarches administratives.

par un site internet ne poserait aucun problème : cela n'a pas été le cas, loin de là. Si la dématérialisation des démarches administratives peut être un incontestable progrès, force est de constater que le numérique n'est pas immédiatement à la portée de tout le monde. S'agissant d'un service public, il doit être conçu afin d'être adapté à tous les publics. Il doit aussi prévoir plus de points d'accueil des personnes peu familières de la pratique informatique, au nombre de 310 actuellement sur l'ensemble du territoire, points animés par des médiateurs qui doivent non seulement être à l'aise avec l'informatique, mais

et de ses missions. Jusqu'à quand ? Nous le saurons très bientôt avec la prochaine réforme de l'organisation territoriale des services de l'État, baptisée « Administration publique 2022 ». Elle doit notamment modifier l'organisation territoriale des services publics, qui prévoit une nouvelle suppression de 50 000 postes de fonctionnaires d'ici à 2022.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera essentiellement sur le programme 216, « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », et spécifiquement sur l'action n° 10, qui concerne la lutte contre la radicalisation. Les occasions de faire un petit point sur ces programmes sont trop rares ; nous allons donc en profiter.

Plus de 4 000 dossiers sont clos. La Commission nationale de l'informatique et des libertés conserve les fiches des « inactifs » pendant cinq ans, mais la place Beauvau précise que « les signalements abusifs ou erronés d'individus qui n'ont jamais été radicalisés ne sont pas conservés dans le fichier ». Ce qui est indéniable, c'est que la menace terroriste demeure. S'y ajoute le problème des « revenants ». On compte aujourd'hui 450 prisonniers jugés pour terrorisme qui seront libérés avant la fin de 2019

avait souligné les défaillances de la politique de lutte contre la radicalisation. Monsieur le ministre, ma question est la suivante : 70 millions d'euros, c'est bien,

En 2010, une fraude massive à l'immatriculation a été découverte, les fraudeurs obtenant extrêmement facilement un numéro d'inscription au répertoire, le NIR- autrement dit, le numéro de sécurité sociale -, sur la base de faux documents. Si vous êtes né à l'étranger, que vous soyez français ou de nationalité étrangère, ce numéro de sécurité sociale vous est attribué manuellement, et il permet donc des fraudes massives sur la base, donc, de faux documents.

radiés. Sur un total de 1,8 million, le compte n'y est pas ! Monsieur le ministre, avez-vous pris des mesures pour faire en sorte que cette fraude massive à l'immatriculation

Monsieur le président, monsieur le ministre,

comprend trois programmes ayant des objectifs diversifiés et d'ampleur inégale : le programme 307, « Administration territoriale » ; le programme 232, « Vie politique, cultuelle et associative » ; le programme 216, « Conduite et pilotage Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », programme « réservoir » qui finance les moyens généraux du ministère de l'intérieur et certaines de ses interventions. La dotation en crédits de cette mission connaît une hausse de 3 % par rapport à la loi de finances pour 2018, soit 83 millions d'euros. Ce n'est pas surprenant. En effet, l'année dernière, les crédits ouverts s'étaient inscrits en forte baisse après le calendrier électoral très dense de l'année 2017 et les mesures de revalorisation salariale alors mises en oeuvre. Je souhaiterais m'attarder surtout sur le programme 307, « Administration territoriale », qui rassemble les moyens des préfectures, hauts-commissariats et sous-préfectures de métropole et d'outre-mer. C'est un programme crucial pour la vie quotidienne des citoyens et des collectivités. Nos préfectures ont connu une réforme importante avec le plan Préfectures nouvelle génération. Mise en oeuvre en 2016, cette réforme a produit ses effets les plus significatifs en 2017 et en 2018. Elle consiste en une réorganisation des services de délivrance de titres- carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire -, afin de moderniser et de simplifier les procédures pour, normalement, améliorer la qualité du service rendu à l'usager. Fondée sur la dématérialisation des procédures, cette réforme a entraîné une réduction très forte des effectifs des préfectures. Celles-ci ont connu la suppression de 1 300 équivalents temps plein entre 2016 et 2018. le réseau préfectoral aura perdu plus de 11 % de ses effectifs en dix ans ; c'est important. l'institution préfectorale, mission régalienne de l'État par excellence et lien direct avec les territoires. Je tiens d'ailleurs ici à saluer la qualité des membres du corps préfectoral. En particulier, je salue le

la reddition d'un forcené qui menaçait de se faire sauter avec une grenade et une ceinture d'explosifs. Cela démontre la variété des missions du préfet. Nous espérons également que la baisse des effectifs ne dégradera pas la qualité et la proximité du service rendu en préfecture. Certains territoires très ruraux ne sont pas équipés d'infrastructures d'accès à internet et se trouvent parfois pénalisés, d'abord en étant éloignés des sous-préfectures où l'on pouvait obtenir la délivrance des titres, puis maintenant en étant dénués de réseau de connexion de qualité pour procéder aux démarches en ligne. La mise en oeuvre de téléprocédures est une bonne chose, mais nous devons veiller à ce qu'elle ne soit pas, pour nos territoires, synonyme d'exclusion. Enfin, nous espérons que cette diminution ne réduira pas les fonctions de conseil et d'ingénierie territoriale auprès des collectivités. L'État, au travers des préfectures, nous le savons bien, est un partenaire crucial des collectivités territoriales. Il faut qu'il conserve les moyens d'accompagner les petites communes. Il est encore trop tôt pour tirer les conséquences de cette réforme du réseau préfectoral ; il faudra en dresser un bilan l'année prochaine avec les services concernés, les collectivités et les usagers. Parmi les plus anciennes institutions de notre État moderne, l'institution préfectorale a toujours fait la preuve de ses capacités d'adaptation au service des Français. Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour ne pas la casser.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'occasion de l'examen des crédits nous pouvons faire quelques variations sur le thème bien connu et éprouvé des réformes structurelles. Les réformes structurelles, tout le monde est pour. Quand on ne porte le fardeau d'être dans la majorité et de soutenir le Gouvernement, on est d'autant plus enclin à réclamer, dans l'abstrait, des réformes structurelles

Cette transformation numérique, je la mets en rapport avec la prochaine phase de la réforme, à savoir la concentration autour de l'équipe préfectorale du pilotage et de l'organisation de l'ensemble des services déconcentrés de l'État,

la mise en commun de toute une série de capacités de service et de systèmes d'information permettra à l'État de devenir plus performant dans sa relation avec les collectivités, mais aussi plus largement avec les citoyens.

et du sens des missions de beaucoup de fonctionnaires de l'État déconcentré. Par comparaison avec les périodes antérieures, l'État est de moins en moins acteur et de plus en plus contrôleur,

société de confiance, il est important de rétablir dans la mission des services déconcentrés et des agents qui les animent une composante « conduite et accompagnement de projets », de soutien

par rapport à 2018, et ce avant tout en raison des prochaines élections européennes. D'ailleurs, sans m'étendre davantage sur le sujet, je soulignerai que le contexte actuel des contrôles des comptes de campagne devrait inviter à interroger les prérogatives de la commission compétente en la matière.

avec des transferts d'emplois d'un autre programme et des investissements comme la mise en oeuvre du réseau radio du futur. On déplore de nouveau ici, malgré les explications qui avaient été fournies, la baisse des moyens du fonds interministériel de prévention de la délinquance. Ces éléments confirment tout simplement le caractère non prioritaire de cette mission et, par conséquent, le choix d'une érosion inexorable des moyens consacrés à l'administration territoriale de l'État. Ce mouvement de repli d'un État de proximité et progressivement « dématérialisé » interroge sur la doctrine territoriale de l'État et les missions du réseau des préfectures.

la numérisation est nécessaire, je m'inscris dans la continuité de ce qui a déjà été dit, pour moderniser notre État, pour l'adapter à une transformation de l'environnement et sécuriser les titres. Cela étant, des difficultés techniques évidentes se sont manifestées dans la mise en oeuvre de cette numérisation, peut-être en raison d'une phase d'expérimentation trop courte, ce qui a non seulement affecté la qualité du service rendu aux citoyens, mais a également terni l'image de l'État. Les nombreux dysfonctionnements informatiques du système d'information des certificats d'immatriculation des véhicules et du site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés, ont conduit à une explosion du nombre d'appels à cette agence, des blocages de dossiers, avec des conséquences fâcheuses, notamment aux niveaux professionnel et personnel, et parfois, je le rappelle, la condamnation de l'État. Des mesures d'adaptation ou correctives ont été apportées, comme le renfort de téléconseillers à l'ANTS, dont le nombre est passé de 48 en 2017 à 175 en 2018, avec l'effet réussi d'avoir impacté l'ambition de réduction budgétaire initiale. La numérisation, c'est très bien ; faire l'impasse sur la fracture numérique, ça l'est légèrement moins. S'il est nécessaire de prendre totalement en compte cette fracture et, pour rappeler ce joli terme

Le Défenseur des droits, qui a fait l'objet de plusieurs milliers de saisines sur le sujet, a dénoncé « les nombreuses atteintes aux droits d'usagers insuffisamment informés en amont de la réforme, trop peu accompagnés une fois celle-ci généralisée et dont les difficultés particulières [d'accès et de maîtrise Pour rappel, 27 % des Français sont toujours sans accès à internet et 33 % maîtrisent peu cet outil. Nous partageons bien entendu les inquiétudes du Défenseur des droits sur ces points. Sa suggestion d'introduire une clause de protection des usagers serait une bonne

La délivrance des titres sécurisés, au coeur du plan Préfectures nouvelle génération, amène à porter un débat de fond sur les missions de l'État dans les territoires. Alors que le PPNG visait à redéployer des emplois sur quelques priorités, les difficultés rencontrées ne l'ont pas permis. La Cour des comptes souligne surtout d'autres missions : la lutte contre le terrorisme, la prévention de la radicalisation et la réforme du droit d'asile. Dans la foulée du rapport Action publique 2022, le Premier ministre a signé deux circulaires pour donner un nouvel élan à la déconcentration, qui soit marqué par une volonté de proximité avec les citoyens par un exercice des missions prioritairement au niveau départemental, voire infradépartemental. Si l'on ne peut s'opposer à cet objectif, l'érosion progressive des moyens de l'administration territoriale laisse songeur quant à sa concrétisation, à plus forte raison avec la suppression annoncée de 50 000 postes de fonctionnaires dans le cadre d'Action publique 2022. En outre, cette affirmation d'une nouvelle déconcentration pose la question de l'adaptation de l'État à l'organisation territoriale et décentralisée de la République, essentiellement sur deux points. Le premier concerne le contrôle de légalité et l'ingénierie territoriale. Le Gouvernement a affirmé sa volonté en matière d'ingénierie territoriale. Je pense, par exemple, à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Dans le même temps, la Cour des comptes estime « souhaitable » la fin de ces missions. En matière de contrôle de légalité, on constate un resserrement du nombre d'actes à transmettre et, surtout, une priorisation des actes à contrôler, inégale entre les préfectures.

Le Premier ministre a demandé aux administrations de « clarifier le rôle de chacun et d'aller au bout du partage des compétences ». Or, pour reprendre une remarque de nos collègues Marie-Françoise Perol-Dumont et Éric Doligé, il y a une tendance quasi naturelle de l'administration déconcentrée à pratiquer l'interventionnisme « touche-à-tout » alors qu'elle n'en a plus les moyens. Cette « clarification des missions » devait reposer, dès la rentrée de septembre 2018, sur une concertation pour une prise de décision à la fin de l'année. Espérons que le climat entre les élus locaux et le Gouvernement se réchauffe et que le mouvement de recentralisation qui est à l'oeuvre depuis quelque temps laisse la place à un recentrage de l'État sur ses missions essentielles. Pour conclure, je rappellerai juste que, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, date de la fondation de l'institution préfectorale, les préfectures et les sous-préfectures étaient avant tout des cuisinières et des drapeaux. En l'état actuel des choses, les cuisinières sont parties, et les drapeaux disparaissent peu à peu de la vie de nos concitoyens, alors même que ceux-ci les réclament comme nous le montre l'actualité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, d'un exercice à l'autre, les crédits de cette mission connaissent d'importantes variations conjoncturelles, rythmées notamment par le calendrier électoral. Ils retracent surtout des évolutions plus profondes, dont l'esprit semble partagé et perpétué par les gouvernements successifs. Car, si les acronymes changent- RGPP, PMMS, RéATE et désormais PAP 2022

Vie politique, cultuelle et associative », doté de 207 millions d'euros, en particulier les crédits de l'action n° 02, Organisation des élections. Ces crédits étant directement corrélés au cycle électoral, leur augmentation de 81 millions d'euros est liée à la perspective des élections européennes de mai prochain. Je profite de cette tribune pour rappeler, comme nous le faisons régulièrement, l'insuffisance de la subvention versée aux communes pour compenser les frais engendrés par l'organisation des élections. Peut-être serons-nous entendus une prochaine fois. Je tiens également à rappeler l'opposition des membres du groupe du RDSE au projet de ne distribuer la propagande électorale que sous sa seule forme dématérialisée. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre de la réforme institutionnelle, étant entendu que « l'illettrisme numérique » devient une véritable question à l'heure du tout-numérique. Les autres actions de ce programme demeurent quant à elles stables, à l'exception de celle qui est destinée à financer la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, en légère diminution et dont les ETP sont gelés. Cette évolution étonne, alors même que les prérogatives et points de vigilance de cette commission ont été accrus dans le cadre de la loi pour la confiance dans la vie politique. Je ne m'attarderai pas sur le programme 216, dont les crédits bénéficient d'une hausse de 3,9 et qui englobe l'administration centrale, la transformation numérique et les affaires immobilières. J'en viens au principal programme de la mission, le programme 307, qui regroupe les moyens alloués au réseau préfectoral. Ses crédits sont en diminution de 2 %, à 1,66 milliard d'euros. La programmation à moyen terme de cette mission confirme un fléchissement continu, bien que, comme l'a rappelé M. le rapporteur spécial, cette trajectoire n'ait pas été totalement respectée. Il en ressort que l'administration territoriale de l'État sera amenée, dans les prochaines années, à se réduire, encore et encore. Vous comprendrez que cela nous interroge, d'autant que, j'y insiste, nous tenons au réseau des préfectures et des sous-préfectures. Quand un nouveau sous-préfet arrive dans mon arrondissement, je lui dis : « Le seul moyen de défendre les sous-préfectures, c'est de faire travailler les sous-préfets. » Sans surprise donc, si les crédits de personnels sur l'ensemble de la mission sont stables, ils sont en diminution de près de 32 millions d'euros dans le programme 307. marque ainsi l'aboutissement du plan Préfectures nouvelle génération, ou PPNG, engagé en 2016. Cette réforme d'envergure repose, en matière de délivrance des titres, sur deux piliers, à savoir la généralisation des procédures dématérialisées et une refonte des modalités de demande et d'instruction, la création d'une cinquantaine de centres d'expertise, les CERT. Dans son rapport pour avis, notre collègue Pierre-Yves Collombat met en lumière certains dysfonctionnements ayant occasionné d'importants délais de délivrance de titres- je pense bien sûr aux cartes grises. Ils ne sont pas nouveaux Il nous interroge aussi sur l'impact de ces réformes sur le service rendu à nos concitoyens et sur la nature même des relations entre le citoyen et l'administration. Dissipons tout malentendu oui, la dématérialisation des procédures constitue un outil privilégié de simplification des démarches pour la majorité des usagers. Elle est une véritable source d'optimisation du service public. Mais on peut s'inquiéter on peut s'inquiéter de l'accès équitable de tous les citoyens aux services de l'État ; je pense notamment aux populations fragiles, celles qui sont frappées par l'illettrisme numérique dont je parlais. Encore faut-il des réseaux pour que les ordinateurs fonctionnent. À cet égard, le Défenseur des droits a relevé, dans sa décision de septembre, une série d'atteintes aux droits des usagers du service public. En attendant, le mouvement de réduction tendancielle des plafonds d'emplois se poursuit. Sur la période 2016-2018, le PPNG se traduit par la restitution de 1 300 ETP. Ces suppressions affectent principalement les échelons départemental et infradépartemental, accentuant le processus de lente dévitalisation de ce réseau et la régionalisation de l'administration.

affichent une hausse de 3 % par rapport à 2018, pour peu, toutefois, qu'ils soient correctement exécutés, leur exécution en 2017 ayant, par exemple, donné lieu à des reports de charges sur 2018. Avec des écarts non négligeables par rapport aux plafonds, la loi de programmation pluriannuelle n'est pas respectée. Le programme 307, « Administration territoriale », couvre le principal vecteur de l'action directe de l'État dans les territoires avec le réseau préfectoral.

Dans le cadre du plan Préfectures nouvelle génération du quinquennat précédent, le Gouvernement s'est efforcé depuis plusieurs années, selon la formule habituelle, de recentrer les missions du réseau préfectoral sur des tâches supposées stratégiques : contrôle de légalité, conseil aux collectivités locales, coordination des politiques. Force est de constater, en pratique, de moins en moins d'accompagnement et de plus en plus de contrôle. D'autres structures devaient alors servir à accueillir les services publics dans les territoires,

En 2019, une baisse de 200 équivalents temps plein est prévue sur l'ensemble de la mission, principalement concentrée sur le programme 307. Cette baisse est inférieure à celle de l'année précédente, mais intervient dans un contexte marqué par un désengagement des préfectures de leur mission de guichet,

Une des conséquences de cette baisse est l'augmentation du nombre de sous-préfectures dotées de moins de 10 emplois, passant de 58 à 76. Il est vrai que le réseau des sous-préfectures s'étiole, étant presque à l'état de quasi-léthargie. Le redéploiement prévu des activités des préfectures vers des tâches plus « stratégiques » s'est heurté à des difficultés, notamment en raison du poids pris par le traitement des demandes de cartes grises, sur lequel a porté, de façon fort opportune, le travail du rapporteur spécial Jacques Genest et qui a parfois conduit au recrutement exceptionnel d'agents non titulaires. Il en est résulté que les emplois redéployables ont été moins importants que prévu, et les futures réductions d'effectifs ne laissent pas présager d'amélioration. On peut s'interroger sur la doctrine territoriale de l'État. Le programme 116, « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », connaît une hausse globale de ses crédits, mais celle-ci est principalement liée à une augmentation des crédits de personnel de l'administration centrale. Il est notable que ce programme est largement un « réservoir » de crédits, qui peuvent être affectés à d'autres missions, ce qui peut engendrer des problèmes d'identification de leur destination finale. Le rapporteur spécial a relevé en commission qu'il s'agissait d'un cas d'information budgétaire « particulièrement défectueuse Je note également que le fonds interministériel de prévention de la délinquance verra ses moyens diminuer par rapport à l'année précédente. Enfin, les dépenses d'action sociale du ministère de l'intérieur s'élèvent à 40 millions

à vous remercier mes propos : je ne réclame pas de réforme structurelle, mais la renaissance d'une organisation territoriale qui a fait la France.

outre le coût financier de cette privatisation de l'ingénierie publique dans un domaine aussi stratégique, les cabinets privés censés suppléer l'absence de l'État sont eux-mêmes largement absents des territoires. Quand ils sont présents, ils manquent souvent du savoir-faire et de l'expérience des ingénieurs des Ponts ou du Génie rural d'antan. Certes, les élus ont fait face, se sont organisés. Les départements et les intercommunalités ont créé des services spécialisés, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, etc. Mais c'est loin d'être le cas partout et les intercommunalités, comme les départements, n'ont aucune obligation en la matière, et toutes ne se sentent pas investies par cette nouvelle mission. Ces solutions restent généralement le fruit d'initiatives locales dont rien ne garantit la pérennité. je ne parle pas des risques de tutelle occulte sur les communes que l'existence de tels organismes peut parfois faire courir. Certes, il arrive, comme je l'ai constaté dans le Doubs que, faute d'alternative départementale ou intercommunale, des préfets maintiennent à la force du poignet un service minimum d'ingénierie en direction des communes rurales. Là encore, il s'agit d'initiatives locales sans garantie de pérennité et qui se limitent essentiellement à l'instruction des dossiers. Ce qui Ce qui inquiète le plus, c'est que ces initiatives ne sont pas vraiment dans l'air du temps libéral, comme se charge de le rappeler la Cour des comptes, qui, comme on le sait, se préoccupe uniquement de bonne gestion et n'assure la promotion d'aucune politique, même libérale. Ainsi, dans son rapport thématique de décembre 2017 relatif aux services déconcentrés de l'État, relève-t-elle : « Bien que la mission d'assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire- ATESAT - ait été supprimée, l'État tend paradoxalement à réinventer des missions de même ordre

une dénonciation au nom de la bonne gestion, qui impose la réduction des services territoriaux de l'État et la chasse aux doublons, avec des missions prétendument à la charge, depuis la loi NOTRe, des départements et des intercommunalités. À la fin du rapport, cependant, la Cour vend la mèche : « Enfin, la conformité de certaines missions de conseil et d'ingénierie territoriale avec le droit européen de la concurrence et des aides de l'État est dans certains cas douteuse, exposant l'État à des risques de contentieux. » Ça, c'est le crime suprême ! L'origine de cette charge, vous le savez, c'est la directive d'orientation de mars 2016, puis la circulaire de juillet 2018 par annonçait qu'il allait enfin se préoccuper d'ingénierie territoriale. Le problème, c'est que, depuis, l'Arlésienne territoriale manque toujours à l'appel, les seules actions observées depuis 2016 étant l'affectation à cette mission prioritaire de 25 postes seulement et un inventaire inachevé des moyens en ingénierie actuellement mobilisables par les préfets. Est-ce donc avoir mauvais esprit de penser que l'annonce de la naissance prochaine d'une agence nationale de la cohésion des territoires, dont on ignore d'ailleurs comment les actions s'articuleront avec celle des préfectures et des organismes de soutien départementaux existants, est un leurre destiné à faire patienter les élus locaux, avant de devenir un moyen de leur faire payer l'addition je ne vous étonnerai pas en vous disant que le groupe CRCE, pour toutes ces raisons et toutes celles que je n'ai pas eu le temps de vous exposer, ne votera pas les crédits de la mission « Administration

une perte d'emploi à hauteur de 1 300 ETP entre 2016 et 2018, dans le cadre du programme Préfectures nouvelle génération. On notera néanmoins une complexité certaine de la lecture du budget réservé à l'administration territoriale. On constatera également une nouvelle baisse des effectifs du réseau préfectoral, avec la perte de 3 357 ETP entre 2007 et 2017. Pour 2019, les suppressions d'emplois prévues touchent principalement l'échelon départemental. La réforme régionale avec la mise en place des grandes régions suscite des inquiétudes, notamment le risque d'éloignement par rapport aux réalités locales. Nous assistons à des fusions, à des jumelages d'arrondissements depuis 2016. Les élus locaux, les habitants restent

Les maisons de l'État et les maisons de services au public permettent de préserver toutefois des accueils de proximité pour le compte des opérateurs et entreprises de services publics publics : La Poste, SNCF, CAF, CPAM, CARSAT, MSA, URSSAF, EDF, GRDF, Pôle emploi, etc. L'administration préfectorale doit faire face à des missions sensibles, notamment l'accueil des étrangers, missions liées également à la sécurité des personnes et des biens,

Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le budget du ministère de l'intérieur compte parmi les premières priorités du Gouvernement. Ses

Peut-être moins souvent commentée ou analysée que les autres crédits dont j'ai la charge, cette mission budgétaire est pourtant à mes yeux- et à vous écouter, à vos yeux aussi -tout à fait fondamentale, et ce pour trois raisons, Elle comprend les crédits de l'administration centrale du ministère, indispensables pour venir en soutien et à l'appui de l'activité opérationnelle de nos forces. Elle abrite les crédits destinés au financement de la vie politique et à l'organisation des élections, qui sont si importants pour la vitalité de notre démocratie. Enfin, elle inclut le budget du réseau des préfectures et sous-préfectures. Je sais, pour avoir été élu local, pendant seize ans, d'une sous-préfecture- la plus grande de mon département, mais elle reste une petite sous-préfecture -, combien ces missions sont fondamentales. C'est tout particulièrement vrai à l'heure où le Premier ministre a souhaité ouvrir le chantier de l'organisation de l'administration territoriale de l'État,

Pour les crédits de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, ce budget est résolument celui de la modernisation au bénéfice de toutes les composantes du ministère, dans une logique de transversalité et de mutualisation des ressources. Ces crédits augmentent de manière significative, à hauteur de 9 %, soit d'un peu plus de 40 Cette augmentation correspond à des projets d'importance, qui sont désormais mûrs pour entrer dans leur phase opérationnelle. Je n'en évoquerai que quelques-uns. Le premier concerne la Tout d'abord, les travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil de 400 postes de travail seront réalisés sur le site de Neuilly en 2019, pour un montant de 20 millions d'euros. Il s'agit d'accompagner la montée en puissance de ce service de renseignement

pour permettre la sécurisation des grands événements à venir, tels que les jeux Olympiques de 2024. Il figurait d'ailleurs parmi les atouts du dossier de candidature de Paris. Le troisième projet d'importance est la mise en place d'un plan de renforcement de la sécurité des applications et systèmes d'information du ministère de l'intérieur.

à l'époque de la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Ce schéma inclut un renfort de 50 personnels au titre des missions nouvelles des préfectures dans le domaine de l'évaluation de la situation des personnes se déclarant mineurs isolés. Pour les personnels de préfecture,

D'une part, il faudra réussir la mise en place de la contribution de l'État à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineurs isolés. C'est un engagement que nous avons pris envers les départements, et nous devons le tenir. D'autre part, il faudra mettre en oeuvre les décisions du comité interministériel à l'intégration,

Le 3 septembre 2018, le Défenseur des droits a rendu un avis dans lequel il fustige la mise en oeuvre de cette réforme : « Ces derniers mois, le Défenseur des droits a traité plusieurs milliers de saisines relatant les difficultés rencontrées avec l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, qui remplace l'accueil auparavant assuré en préfecture ou sous-préfecture par des démarches en ligne.

moyens, votre demande me paraît satisfaite : en 2018, 90 agents supplémentaires ont été affectés aux centres d'instruction des demandes d'usagers, situés à Amiens, à Charleville-Mézières et à la préfecture de police. En outre, les effectifs de l'ANTS dédiés à la prise en charge directe des usagers ont été triplés. Ils ont ainsi été portés à 180 personnes.